associés ; Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont le Sénat est saisi en application de l’article 47 1, alinéa 2, de la Constitution

est à Mme la ministre. En application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande la réserve de l’article 8, sans les amendements portant article additionnel après cet article, afin que celui ci soit examiné juste avant l’article 11.

En cohérence avec les recommandations du rapport, cet amendement tend donc à supprimer les mécanismes d’exonérations de cotisations sociales dits bandeau famille et bandeau maladie uniquement pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 Smic.

En effet, retenir comme plafond sa valeur au 1 janvier 2024 aurait pour effet d’alourdir le coût du travail pour les entreprises. Par principe, je suis opposé à toute nouvelle augmentation du coût du travail. à rétablir un niveau de chômage correct depuis plusieurs années : voulons nous vraiment effectuer un retour en arrière ?

Il s’agit bien souvent de sociétés qui œuvrent dans des secteurs très concurrentiels à faible marge, comme celui du transport de marchandises. Le texte qui nous est présenté acte la suppression de la prise en compte des déductions au titre de frais professionnels, calculées forfaitairement, pour le calcul de la réduction générale dégressive, qui plus est avec une rétroactivité au 1 janvier 2024, ce qui aurait un effet dévastateur pour l’ensemble des secteurs

préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression. La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour le personnel roulant, tels que l’augmentation de leur salaire net. En permettant En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d’autant plus cruciale dans le secteur du transport routier que les frais professionnels sont particulièrement élevés : frais de déplacement, hébergement, repas… En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, ce financièrement les salariés qui se déplacent au quotidien et rend la profession plus viable économiquement. Dans le contexte socio économique actuel, où le secteur des transports connaît un niveau de défaillances inédit, une telle rétroactivité viendrait mettre à mal la santé financière d’entreprises déjà en difficulté. La

le coût du travail sur les bas salaires. En 2023, la Commission des comptes de la sécurité sociale évaluait le coût des exonérations de cotisations sociales sociales à 89 milliards d’euros, soit près de 3 points de PIB, dont 2,9 milliards n’étaient pas compensés par le budget de l’État. Dans le total de ces exonérations, le bandeau maladie représentait un coût de 25 milliards

consolidées, selon les critères européens. Pour les comptes sociaux, une remise en cause des bandeaux à partir de deux fois le Smic réduirait les exonérations et donc la dépense pour l’État. Ces exonérations

du Conseil d’analyse économique, si les baisses de cotisations sociales sur les bas salaires ont pu avoir des effets sur l’emploi, elles n’en ont plus au delà du seuil de 1,6 Smic. Même les économistes mandatés par le Gouvernement, MM. Bozio et Wasmer, ne relèvent pas d’effet sur

ne cesse de peser sur le budget de l’État et les comptes de la sécurité sociale, les divers gouvernements s’obstinent à ne pas remettre en cause des politiques d’exonérations qui sont sans effet au delà d’une certaine limite. Placer un point de sortie à 2 Smic serait une stratégie bien meilleure que la cure d’austérité

à la direction que souhaitait imprimer l’ancien Premier ministre. Par ailleurs, selon une étude du Conseil d’analyse économique de 2019,

nous semblent trop brutales pour nos entreprises. Je pense à l’amendement n° 122 de Mme la rapporteure générale. En fixant le seuil de sortie de la réduction générale à deux fois le niveau du Smic, nous ferions peser sur nos entreprises un effort plus élevé de 500 millions d’euros que celui résultant de la proposition du Gouvernement, avec un impact néfaste en termes de compétitivité et d’emploi. Il est essentiel de préserver le tissu industriel de notre pays.

de décider qu’une entreprise est plus ou moins polluante. Cependant, des entreprises, y compris dans le secteur pétrochimique, peuvent tout à fait s’engager dans

Par cet amendement, je propose de mettre en place un comité de suivi. Nous avons eu l’occasion d’en parler, madame la ministre, et je pense que vous êtes assez favorable à cette perspective.

Depuis trente ans que les entreprises bénéficient d’allégements de cotisations sociales, dont le montant atteindra 80 milliards d’euros en 2025, une évaluation de leur efficacité ne serait pas du luxe. En réalité, les comités d’évaluation des aides publiques aux entreprises ont déjà existé. Ainsi, après sa création, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi a fait l’objet, chaque année, d’un rapport public d’évaluation. ont d’ailleurs tous démontré un écart entre l’efficacité du dispositif et le coût pour la sécurité sociale. C’est pourquoi nous souhaitons que vous puissiez créer des comités de suivi régionaux,

Madame la sénatrice, votre amendement vise à reporter d’un an, soit au 1 janvier 2026, l’extension du champ d’application du bulletin officiel de la sécurité sociale au régime agricole. Il est vrai que les premières rubriques ont d’abord porté sur des dispositifs propres aux salariés du régime général. Toutefois, les salariés agricoles et leurs employeurs ont également le droit de disposer d’une information claire et opposable sur leurs cotisations et les contributions sociales. Les spécificités propres au régime agricole seront bien évidemment prises en compte. Des discussions entre le ministère de l’agriculture et la direction de la sécurité sociale, qui est responsable de la publication du bulletin, sont déjà organisées pour publier dès l’année prochaine des contenus spécifiques à ces travailleurs. Pour ces différentes raisons, je vous demande de retirer cet amendement ; à défaut, j’y serai

Lodéom, des effets indirects de la refonte des allégements généraux prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Aujourd’hui, toute modification du régime général impacte automatiquement la Lodéom en raison de l’imbrication des textes législatifs. l’amendement vise à geler les paramètres actuels du régime Lodéom afin de neutraliser les ajustements envisagés, tels que la fixation par décret du Smic de référence, la suppression de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l’intégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette des allégements. qu’elles aient un effet rétroactif au 1 janvier 2024, risquent d’entraîner une hausse du coût du travail et des prix, aggravant le coût de la vie dans des territoires déjà fragiles. En maintenant les paramètres actuels, nous protégeons la dynamique d’emploi favorable observée depuis trois ans en outre mer et évitons une pression supplémentaire sur des secteurs essentiels, comme le transport et la construction. Enfin, les organisations économiques ultramarines se disent prêtes à engager des discussions en 2025, sur la base d’analyses d’impact et d’évaluations précises, pour envisager des évolutions adaptées et concertées. Il est de notre devoir de préserver le dispositif de la Lodéom, qui est vital pour nos territoires ultramarins. La parole

de calcul. Mais l’idée qu’il ne consulte pas les parlementaires sur des enjeux aussi cruciaux ne nous convient pas. Les collègues ultramarins se sont exprimés

Cet amendement est le même que celui de Mme la rapporteure générale. Il s’agit de geler les paramètres actuellement applicables au régime d’exonération de charges sociales patronales spécifique aux outre mer. Il ne saurait être question d’inscrire dans nos actuels débats budgétaires des mesures non concertées, car cela casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre mer et renchérirait inexorablement le coût du travail avec des répercussions inévitables sur les prix, donc sur le coût de la vie.

et en maintenant la déduction forfaitaire spécifique pour certains secteurs clés, comme la construction et le transport. Il tend également à exclure les entreprises ultramarines de la réduction progressive des exonérations de cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales, ainsi que de l’abaissement du taux maximal d’exonération pour les salaires proches du Smic. En outre, il a pour objet de s’opposer à toute modification de ces mesures par ordonnance sans consultation parlementaire. De fait, de telles réformes aggraveraient les difficultés de secteurs déjà fragiles, comme le transport, et augmenteraient le poids des prélèvements sociaux, ce qui impacterait fortement les entreprises dans un contexte marqué par un chômage élevé et un coût du travail important.

Comme le ministre des outre mer, François Noël Buffet, l’a indiqué lors de son audition devant la délégation sénatoriale aux outre mer le 7 novembre dernier, toute modification du régime d’exonération des cotisations sociales doit faire l’objet d’une évaluation et d’une concertation approfondies,

Ce projet de réforme, tel qu’il est envisagé par le Gouvernement, risque d’avoir d’importantes répercussions sur le tissu économique, déjà très fragile, de nos territoires. Les inquiétudes sont vives, et l’ensemble des acteurs sont vent debout face à cette menace. Bien que je salue l’amendement de la commission, le recours aux ordonnances, même dans un champ d’habilitation

En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 6 du PLFSS, les entreprises situées en outre mer qui déclarent des salariés sous le régime des allégements généraux seront, par définition, impactées de la même manière que les entreprises hexagonales par ce projet de réforme dès le 1 janvier 2025.

Dans un contexte de chômage endémique et de grande précarité, l’adoption, en l’état, de ces deux dispositions constitue une menace très forte sur la pérennité du tissu économique existant, donc sur les emplois en outre mer. chers collègues, le sujet est grave. J’ai été alerté sur les risques de l’application de cet article par plusieurs fédérations d’entreprises, en particulier par M. Laval, référent martiniquais de la Fédération des entreprises de services à la personne et dirigeant des structures Zen à domicile et Abivi, qui emploient 189 salariés intervenant auprès de 511 familles sur mon territoire. Cet amendement de bon sens et de prudence vise à protéger l’emploi en outre mer. La parole

réforme. Je ne reviendrai pas sur les propos que j’ai tenus en discussion générale, mais je tiens à alerter sur ces économies en trompe l’œil. Je rappelle que Saint Barthélemy bénéficie d’un dispositif spécifique, qui a été introduit pour lui permettre de faire face à la concurrence. à la concurrence. Encore aujourd’hui, devant la commission des lois, le ministre des outre mer a indiqué son souhait de se projeter, avec notamment des documents stratégiques par collectivité. Je souscris à cette position et considère que les exonérations devront faire partie de la définition d’une vision stratégique.

En effet, dans les collectivités d’outre mer, la majorité des entreprises sont des TPE ou des PME de moins de onze salariés. Celles ci emploient des personnes implantées localement et sont des piliers des économies locales ultramarines. La réforme du régime des allégements généraux de cotisations sociales patronales aurait des conséquences délétères pour les salariés et la pérennité des entreprises, selon l’étude d’impact fournie par le Gouvernement. Les économies ultramarines, déjà fragiles, ne pourraient pas supporter ce nouveau choc. Les défaillances d’entreprises ne cessent de croître : à titre d’exemple, elles ont L’étude d’impact du gouvernement précise bien que cette réforme impacterait le coût du travail. Les victimes en seraient à la fois les entreprises et les salariés. L’adoption de cet amendement est donc nécessaire pour protéger les entreprises et les économies ultramarines, qui ne peuvent absorber un nouveau choc.

l’amendement n° 668. Cet amendement a pour objet de ne pas intégrer la prime de partage de la valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allégements et de maintenir en l’état le dispositif de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les entreprises des territoires ultramarins. Il tend également à exclure ces dernières de l’extinction progressive annoncée des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales, de l’abaissement progressif de deux points, dès 2025, puis de quatre points, dès 2026, du taux maximal d’exonération au niveau du Smic et, enfin, de réfuter le principe d’une habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales applicables aux outre mer. Pour les raisons que nous avons déjà évoquées, il n’est pas raisonnable d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, sans le moindre contrôle préalable du Parlement,

tiens à réaffirmer que l’intention du Gouvernement est bien de neutraliser les effets de certaines de ces dispositions de manière à maintenir un avantage

par ordonnances et c’est pourquoi geler les paramètres de la Lodéom au 29 décembre 2020 de manière définitive n’est pas souhaitable.

aux députés et sénateurs intéressés par la question, indiquent que ce dispositif, comme les allégements généraux de droit commun, n’incite pas les employeurs à augmenter les salaires, lorsque ceux ci sont au niveau

Vous proposez également que la diminution des points de sortie des réductions proportionnelles de cotisations maladie et famille au 1 janvier 2025 ne soit pas applicable aux employeurs qui bénéficient par ailleurs de dispositifs d’exonération spécifique. spécifique. À mon sens, de telles dispositions ne sont pas justifiées. Actuellement, tous les employeurs bénéficient dans les mêmes conditions de dispositifs de réduction générale des cotisations sociales. Ce sont les réductions dégressives qui, quant à elles, sont parfois différenciées selon les employeurs. Rien ne justifie d’introduire une différence dans le cadre d’un dispositif général au motif que l’on bénéficierait par ailleurs d’un dispositif spécifique. En outre, cela emporterait des conséquences opérationnelles lourdes

Demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes sans qualification, etc. : 64 % d’entre eux connaissent une sortie positive et retrouvent le chemin de l’emploi. Mes chers

codifiée dans aucun texte, expliquant que des entreprises bénéficient d’un régime d’allégement antérieur à une certaine loi. Il conviendrait plutôt d’insérer un dispositif spécifique

ont été mises en place en faveur des employeurs implantés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint Barthélemy et à Saint Martin. Il s’agit du dispositif Lodéom. Jusqu’à ce

Merci,

environnementale, salariale et de plan de licenciement. Par ailleurs, en rétablissant les cotisations patronales à la branche famille, nous pourrions financer un véritable service public de la petite enfance. En ce mardi 19 novembre, nous avons évidemment

construction, non générateur de droits et exempté de cotisations. Selon la Cour des comptes, l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur ne sont pas compensés pour les comptes de la sécurité sociale, même après prise en compte des forfaits sociaux. ces forfaits sociaux ont récemment été abaissés pour nombre de ces dispositifs, de sorte que l’ensemble contribue de plus en plus à grever les recettes de la sécurité sociale. Au total, les pertes de recettes relatives aux compléments de salaires exonérés et non compensés

et médico sociaux (ESSMS) associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019, de cet abattement de charges pérenne,

d’autofinancement suffisante. Cette situation s’est fortement aggravée entre 2022 et 2024, l’écart entre l’augmentation des charges liée à l’inflation

Dans le secteur sanitaire, cette différence entre le secteur public et le secteur privé est compensée par les tarifs. Une telle différence de traitement pénalise toutefois les établissements sociaux et médico sociaux publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes et il est inéquitable de les surtaxer.

et publics, dans l’objectif de tendre vers la neutralisation d’une éventuelle différence de traitement socio fiscale entre ces établissements. En tout état de cause, je partage avec vous l’objectif de redonner des marges de manœuvre financières aux établissements du secteur public et d’assurer une équité entre les statuts

prévoit déjà que les niches sociales ne peuvent excéder 14 % des recettes des régimes obligatoires de base, ce qui implique en pratique de respecter une règle de gage de ce type.

démontrant l’explosion du manque à gagner pour les comptes sociaux des exemptions provoquées entre autres par l’abaissement des forfaits sociaux et exemptions non compensées. La Cour des comptes pointait ainsi la baisse importante du rendement des taxes compensatoires, qui est passé de 43,5 en 2018 à 35,6 % en 2023, du fait entre autres des nombreux abaissements des forfaits sociaux, dont celui ci. Cet abaissement a eu un effet d’aubaine, selon la Cour, puisque « parmi parmi l’ensemble des dispositifs exemptés, les stock options et les attributions gratuites d’actions ont connu la progression la plus forte, +36 % par an entre 2018 et 2023, compte tenu de leur régime dérogatoire favorable ». En conséquence, la Cour recommandait que, au minimum, la contribution de l’employeur soit rétablie à 30 %. Cette mesure peut être chiffrée à près de 400 millions d’euros de recettes supplémentaires pour la sécurité

selon un mécanisme de rémunération complémentaire qui vise à motiver et à fidéliser certains salariés. Jusqu’en 2015, le taux de contribution patronale applicable aux attributions gratuites d’action était de 30 %. La loi du 6 août 2015 pour la croissance,

ont tantôt augmenté, tantôt réduit le taux de contribution patronale sur les actions gratuites. La question primordiale est, selon nous, de savoir qui bénéficie d’actions gratuites et pour quelle utilité.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de relever le taux de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites de 20 % à 30 %. Cette hausse de dix points ne remettrait pas en cause la distribution d’actions gratuites, mais permettrait de dégager

« part extrêmement restreinte ». Il permet une plus forte implication des bénéficiaires et favorise le développement de l’entreprise, objectif auquel nous sommes tous attachés.

notamment une recommandation concernant la mise en cohérence de la fiscalité et du traitement social des dispositifs d’actionnariat salarié avec le système d’attribution d’actions

charge des arrêts maladie. Nous proposons donc de rétablir les cotisations sociales sur la prime de partage de la valeur pour inciter les employeurs à privilégier des augmentations de salaire durables qui bénéficieront à la fois aux salariés et au financement de la sécurité sociale.

ne semble pas souhaitable. Cet instrument a permis de soutenir le pouvoir d’achat des salariés durant la période d’inflation récente et offre, de plus, une flexibilité aux TPE et PME de notre territoire qui voient leur activité perturbée par le contexte économique. Par ailleurs, la PPV a fait l’objet d’un accord national interprofessionnel, signé par l’ensemble des partenaires sociaux représentatifs, à l’exception de la CGT. Revenir sur ce point serait trahir l’engagement de transposition de cet accord

En effet, dans le cadre de leur développement, les intercommunalités, pour mutualiser significativement leurs coûts, confient de plus en plus souvent aux syndicats mixtes fermés la gestion des services d’aide et d’accompagnement à domicile et participent ainsi aux politiques tant nationales que départementales de maintien à domicile et d’action sociale. Pour autant, les syndicats mixtes fermés ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d’un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté. Cette différence de traitement est d’autant plus incompréhensible que les CIAS bénéficient de cette exonération. Une régularisation permettrait par ailleurs de lutter efficacement

a pour objet les interventions effectuées au sein des sociétés de téléconsultation. Il vise à compenser le montant des cotisations sociales des médecins salariés en secteur 1 pour l’aligner sur celui des médecins libéraux par le truchement d’une exonération. C’est aussi une mesure d’égalité. En effet, l’ensemble des structures qui salarient ces médecins exerçant en secteur 1 bénéficient de cette compensation. Cette mesure permettra d’encourager la prise en charge en secteur 1 par les médecins salariés des sociétés de téléconsultation.

qui concerne 7 millions de salariés et 600 000 agents publics. Une telle mesure aurait un effet direct sur le salaire net des salariés concernés.

pas pour répondre à cette crise. Nous proposons d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur. Cette disposition bénéficierait directement aux salariés, ainsi qu’aux employeurs, et aurait donc un effet immédiat sur l’attractivité des métiers de l’aide

Il convient, selon moi, d’en rester aux principes applicables actuellement, car ils correspondent à une réalité objective : la mise à disposition d’un véhicule pour un usage strictement professionnel ne constitue pas un avantage en nature, à la différence d’une mise à disposition permettant un usage personnel.

générale des finances de 2016 souligne la spécificité des besoins des travailleurs handicapés. Ce rapport témoigne d’un vieillissement de la population, d’une fatigabilité accrue,

par voie réglementaire pour limiter ce risque. Nous visons ainsi une plus grande mutualisation du coût des maladies professionnelles à effet différé, afin de lever un frein supplémentaire à l’emploi des salariés en situation de handicap.

Ainsi, dans les entreprises adaptées, les salariés en situation de handicap sont ils plus âgés et vulnérables que dans les entreprises classiques. Cette situation affecte naturellement le taux de cotisation AT MP de ces entreprises, et c’est pourquoi cet amendement vise à ce que les modalités de calcul de ce taux puissent être modifiées. objectif est de parvenir à un taux mutualisé qui serait quasiment indolore pour les entreprises et qui soulagerait financièrement les entreprises employant de nombreux salariés en situation de handicap.

terrain, et ne semble pas justifiée, notamment pour les maladies professionnelles dont l’effet est différé. Renforcer la mutualisation du risque entre les employeurs pour les maladies professionnelles à effet différé subies par les bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé pourrait donc lever un frein à l’emploi des personnes en situation de handicap. Une mesure identique a été prévue, lors de la réforme des retraites – un mauvais souvenir pour certains,

qui prévoit une mutualisation, entre les entreprises, des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps. Les deux amendements visent à préciser que ledit dispositif s’applique également aux travailleurs handicapés.